madame la présidente,

vise à mettre en valeur dans la constitution des communautés professionnelles territoriales de santé, ou CPTS, les intervenants de premier recours que sont les acteurs du domicile ou les structures ambulatoires intervenant dans le champ de l'enfance en situation de handicap. Outre les deux catégories de structures permettant de lier les professionnels de santé libéraux avec des structures d'intervention précoce, sont donc visés par cet amendement les services d'aide et d'accompagnement à domicile- Saad les services de soins infirmiers à domicile- Ssiad -et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile- Spasad -pour personnes âgées et personnes en situation de handicap. Sont également visés les services nécessitant une orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, tels que les services d'éducation spéciale dans le champ de l'enfance, les services d'accompagnement à la vie sociale et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Si l'ensemble des établissements et services médico-sociaux sont ciblés par le projet de loi actuel, il semble important, dans le cadre de la promotion d'une société plus inclusive pour les personnes fragiles ou non encore diagnostiquées dans le champ de l'enfance en situation de handicap, de mieux faire coopérer les professionnels de santé du premier recours avec les structures de ville ou les services intervenant au domicile de ces personnes, afin de renforcer le soin de premier recours et de mieux positionner les interventions des services à domicile ou d'accompagnement spécialisé sur des missions de prévention. Quel

de la commission ? Le code de la santé publique donne une définition large de la CPTS, qui peut réunir des professionnels, mais aussi « des acteurs médico-sociaux et sociaux concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé

En créant ce statut, la CPTS se dote d'une personne spécialisée pour coordonner tous les professionnels de santé du territoire. Cela permet une plus grande stabilité et le recrutement de personnes compétentes, disposant de moyens d'actions pour piloter des projets, notamment des projets de long terme.

cet amendement tend à inscrire, dans le code de la santé publique, la possibilité pour les établissements de santé de participer aux communautés professionnelles territoriales de santé. Cette association se fera sur l'initiative de la CPTS, si elle le souhaite.

est à Mme Annie Delmont-Koropoulis. Il ne paraît pas acceptable que les professionnels de santé et médico-sociaux ne soient pas libres de déterminer le périmètre de leur CPTS, ni que leur projet de santé soit soumis à approbation. Soumettre à approbation administrative une organisation de soins ambulatoires démontre une volonté d'hyperadministration, peu cohérente avec d'autres dispositions de ce projet de loi. Pour que notre système de santé se porte mieux et que le maillage territorial puisse s'opérer dans de bonnes conditions pour les professionnels de santé, il est essentiel de faire confiance aux acteurs de terrain. Ces derniers travaillent déjà ensemble sur leur capacité à se regrouper à une échelle pertinente et à proposer des projets cohérents avec les projets territoriaux de santé. Cet amendement a donc pour objet de supprimer la surcouche administrative administrative prévue à l'alinéa 17 de l'article 7, afin de renforcer la confiance accordée aux acteurs de terrain : ils sont les plus à même d'apporter des solutions organisationnelles pérennes pour améliorer l'accès aux soins. Quel est l'avis de la commission ?

en approbation implicite, sauf opposition de l'ARS. Une telle rédaction me semble marquer plus clairement l'esprit de confiance et de souplesse que je souhaite insuffler dans ce projet de loi. Au-delà, il ne me semble pas souhaitable de supprimer totalement le droit de regard de l'ARS sur le projet de santé des CPTS.

CPTS. Si l'on ambitionne de favoriser le développement d'un exercice coordonné, la responsabilité de ce diagnostic doit être étendue aux équipes de soins spécialisés, qui jouent un rôle important, avec l'augmentation des maladies chroniques. Ces équipes, constituées autour de médecins spécialistes d'une ou plusieurs branches, sont en mesure d'apporter des compétences nécessaires

prévus à l'alinéa 20 de l'article 7, de revoir, avec l'accord de tous les partenaires, des modalités de financements plus adaptées aux spécificités de ces territoires. Dans le prolongement des préconisations du rapport de Jean-Marc Aubert sur le financement du système de soins dans les départements d'outre-mer, cet amendement vise à proposer de nouveaux modes de financement pour les groupements plus proches de la réalité de ces établissements et fondés sur une contractualisation entre les différents partenaires de chaque territoire. En effet, les établissements de santé des outre-mer connaissent, dans leur majorité, des difficultés financières que les pouvoirs publics pallient depuis de nombreuses années, sans revoir les modes de financement et les coûts induits par l'éloignement. Ainsi, les coefficients géographiques appliqués aux tarifs en outre-mer et les coûts des évacuations sanitaires sont souvent sous-estimés et doivent, de l'avis de tous, être révisés, tant leurs calculs sont peu transparents et, donc, inadaptés aux enjeux de chaque département ultramarin. Des difficultés de mobilité et la mise aux normes de ces établissements sont autant de problématiques qui impactent lourdement leurs trésoreries déjà fragiles. Il s'agit par cet amendement de permettre, en accord avec les ARS et dans le cadre des contrats territoriaux de santé,

lors de ses déplacements en outre-mer, en 2016 à La Réunion, puis en 2018 en Guadeloupe. Toutefois, la commission ne pense pas que ce soit le rôle des contrats territoriaux de santé que de prévoir des modalités de financement dérogatoires de l'hôpital dans les outre-mer. Ces contrats sont en effet conclus sur la base des projets des CPTS ou des futurs PTS. La commission demande donc le retrait de cet amendement

au niveau national et je préfère que nous travaillions ainsi : sur l'ensemble du modèle économique des établissements de santé et dans le cadre approprié, actuellement en cours de concertation. Avis défavorable,

Déjà synonymes d'angoisse, ces services se sont tristement illustrés par des faits divers, ayant malheureusement entraîné la mort de patients, ainsi que par des dérapages budgétaires. Cet amendement traduit une recommandation de la Cour des comptes afin de résoudre, en partie, un des problèmes majeurs : le temps d'attente pour la prise en charge.

et d'autres types d'actes plus lourds qui nécessitent son attention. Le décret permettra de consulter en amont l'ensemble des ordres concernés, afin de déterminer une liste acceptée par l'ensemble des professionnels de santé. professionnels de santé. Quel est l'avis de la commission ? L'objectif est partagé : il s'agit d'améliorer les conditions de prise en charge des patients et de libérer du temps médical en assurant des délégations d'actes vers les infirmiers. ces possibilités sont déjà prévues : dans le cadre des infirmiers de pratique avancée ou encore des protocoles de coopération, dont nous souhaitons la montée en puissance. Les services d'urgence seraient en effet un domaine dans lequel de nouvelles formes de délégations d'actes pourraient se développer. Les outils existant déjà, l'amendement est satisfait.

à l'article 19 de ce projet de loi, un cadre considérablement assoupli va vous être proposé pour accélérer et simplifier l'approbation de protocoles de coopération entre les professionnels.

au niveau départemental, sur l'organisation territoriale des soins, de façon à assurer la bonne coordination de l'action des collectivités territoriales et des agences régionales de santé. Il prévoit également la possibilité, pour les élus, d'entendre le directeur général de l'agence régionale de santé sur un point qu'ils souhaiteraient inscrire à l'ordre du jour. En effet, une coordination entre les agences régionales de santé et les collectivités territoriales est déjà à l'oeuvre au niveau régional, au sein des commissions de coordination des politiques publiques. Il s'agit, par cet amendement, de prévoir un mécanisme complémentaire au niveau départemental.

et les nombreux facteurs qui le déterminent- environnements, professionnels de santé, établissements et services de soins et d'accompagnement, etc. -est indispensable dans une perspective d'aide à la décision, d'ingénierie et de mise en place de politiques publiques. Malheureusement, ces données ne sont pas toujours accessibles aux décideurs publics et élus, alors même qu'elles permettraient de mettre en lumière certaines problématiques. C'est notamment le cas dans certains territoires dépourvus d'observatoires de santé, comme dans le Nord et le Pas-de-Calais. Face à ce constat, il nous semble pertinent que l'ARS partage les données dont elle dispose en la matière et en fasse une présentation au moins annuelle aux élus du territoire concerné. C'est ce que mon groupe propose au travers de cet amendement.

en adaptant l'offre aux besoins locaux et contribuent à la maîtrise de l'Objectif national de dépenses d'assurance maladie dans le respect de la mission fixée par le législateur aux ARS. Des instances de concertation ont été mises en place pour consulter les acteurs du système de santé que sont les élus, les professionnels de santé et les usagers, parmi lesquels les conseils de surveillance des ARS, la conférence régionale de santé et de l'autonomie et les conseils territoriaux de santé. Mais aucun dispositif n'est prévu à l'heure actuelle pour permettre aux directeurs généraux des ARS de présenter leur politique locale de santé aux élus du territoire. Dans la continuité de l'engagement de Mme la ministre nationale lors de la séance de questions au Gouvernement du 12 mars dernier, il est important que les ARS fassent un travail commun avec les élus locaux, mais aussi les professionnels de santé, les citoyens et les usagers du territoire. Cet amendement prévoit que le directeur général de l'agence régionale de santé leur présente régulièrement le bilan de la mise en oeuvre de la politique de santé sur le territoire concerné, notamment en matière d'accès aux soins et d'évolution de l'offre de santé. Il s'agit de permettre en outre au directeur de l'ARS, ou à son représentant, de convier les associations agréées en matière de santé,

Mme Laurence Cohen. Notre amendement vise à réintroduire une disposition supprimée par la commission des affaires sociales, à savoir la présence des parlementaires du département

et des maires s'opposerait à la présence des parlementaires du département. Les PRS sont une mine d'informations sur la réalité sociale et sanitaire de nos départements. De plus, ils entérinent les politiques publiques locales en matière de santé pour quatre ans, que ce soit en matière de lutte contre les inégalités sociales et territoriales d'accès aux soins, de prévention, de vieillissement de la population, de santé environnementale. Autant de sujets qui méritent que nous assistions à la présentation qui, je vous le rappelle, mes chers collègues, donne lieu à un débat. Permettez-moi d'illustrer mon propos par un exemple. En Île-de-France, le PRS 2, adopté voilà près d'un an, prévoyait de maintenir deux hôpitaux en capacité de réaliser des greffes hépatiques dans le Val-de-Marne. Malheureusement, le directeur de l'AP-HP a décidé de n'en garder qu'un. Il serait

des décisions que l'on peut mieux défendre l'intérêt des patients et des professionnels. Telle est, en tout cas, notre conception de la démocratie sanitaire.

Cet amendement n° 545 rectifié évoque mieux l'idée d'une réunion de concertation, alors que la rédaction issue de l'Assemblée nationale évoquait davantage celle d'une présentation par l'ARS sous la forme d'une information « descendante

L'amendement n° 699 traduit une demande légitime de disposer de données de santé publique, mais celles-ci sont déjà disponibles par ailleurs. Sa rédaction est du reste incompatible avec celle de l'amendement n° 545 rectifié. Avis défavorable. Enfin, la

face au manque de médecins généralistes dans les territoires, il est de plus en plus difficile pour nos concitoyens de trouver un médecin traitant, qui, on le sait, est la pierre angulaire de notre système de santé. Les patients ayant un médecin traitant ont la possibilité, d'une part, d'être mieux soignés grâce à un suivi régulier adapté à leur état de santé, et, d'autre part, d'être mieux remboursés, notamment lorsque le médecin traitant est consulté avant orientation vers un autre professionnel de santé. Pour tenter de répondre au problème, le code de la sécurité sociale permet aux médecins d'une même spécialité au sein d'un même cabinet médical ou d'un même centre de santé d'être conjointement désignés médecins traitants. Si les projets de regroupement de cabinets médicaux ou de création de centres de santé se développent, cette avancée reste insuffisante et trop restrictive. Aussi, l'amendement que je vous propose d'adopter a pour but de permettre aux médecins d'être désignés conjointement médecins traitants dès lors qu'ils participent à une même communauté professionnelle territoriale de santé. Les CPTS ont pour objectif de regrouper les professionnels de santé au sein d'un même territoire autour d'un projet médical et médico-social commun. Si la proposition que je vous fais n'est pas un remède miracle,

la possibilité pour des médecins exerçant la même spécialité au sein d'un cabinet médical ou dans un centre de santé d'être conjointement désignés médecins traitants. Il paraît pertinent d'étendre cette faculté aux médecins exerçant dans le cadre d'un

d'un amendement que nous avions adopté en commission d'aménagement du territoire et traitant de l'organisation des systèmes de garde pour les professionnels des CPTS, dans le cadre des négociations conventionnelles avec l'assurance maladie, à ceci près que nous avions introduit l'échelle des bassins de vie. Cette mesure est essentielle pour garantir à chacun de nos concitoyens un accès aux soins, au plus proche de chez eux. Il est en effet intolérable qu'en France des gens ne trouvent pas de médecin de garde à proximité de leur domicile.

pour déterminer des modes de financement pérennes des CPTS et préciser leurs missions en accord avec les professionnels de santé concernés. D'après les indications du directeur général de la CNAM, l'accès à des plages de soins non programmés ferait ainsi partie des missions socles de ces CPTS, conditionnant l'accès aux financements prévus. Il n'est donc pas opportun

hospitalier et en créant un statut d'assistant orienté vers l'activité libérale. Nous essayons d'apporter une autre réponse pour résoudre les problèmes de démographie médicale. Ce nouveau dispositif orienté vers l'activité libérale serait proposé aux jeunes médecins thésés, et viendrait en appui des professionnels de santé, quel que soit leur modèle de regroupement. Il produirait des effets à court terme sur la professionnalisation et, surtout, l'installation des médecins. Quel

En effet, l'ouverture d'une première officine est autorisée lorsque le nombre d'habitants recensés est au moins égal à 2 500. En revanche, pour pouvoir en ouvrir une de plus, l'autorisation est délivrée par tranche supplémentaire de 4 500 habitants. Ce second seuil est trop élevé et empêche ainsi, sur de nombreuses collectivités, l'installation d'une deuxième pharmacie, alors que les besoins liés à la desserte en médicaments sont bien présents. Dans plusieurs communes de l'Essonne, ce seuil empêche l'implantation d'une officine supplémentaire. Pourtant, de nombreux patients de communes voisines viennent dans ces dernières se fournir en médicaments. Une seule pharmacie est donc loin d'être suffisante. C'est pourquoi, par cet amendement, nous proposons d'établir un seuil raisonnable pour l'ouverture d'une deuxième officine : 2 500 habitants au lieu de 4 500. Toutefois, la tranche supplémentaire de 4 500 habitants pour l'ouverture d'une pharmacie de plus reste inchangée. Par ailleurs, les conditions démographiques sont appréciées pour une durée au moins égale à deux ans. Là aussi, ce critère est trop contraignant, notamment lorsque l'évolution démographique est avérée ou prévisible. Cet amendement vise à réduire ce délai à un an.

à l'installation d'une nouvelle officine sur le territoire d'une commune, du fait des seuils démographiques. Toutefois, le maillage officinal est aujourd'hui excellent. Alors qu'une ordonnance parue en janvier 2018 a adapté les conditions de création des officines, il ne paraît pas à la commission opportun de revenir sur les équilibres actuels sans associer la profession,

Une telle pratique pose de sérieuses difficultés, en particulier quand les besoins d'approvisionnement et d'accès des populations, présents et à venir, ne sont plus satisfaits. Cette pratique s'est illustrée à au moins deux reprises dans le département de l'Essonne. Dans le premier cas, une commune a vu sa seconde pharmacie fermer après que les propriétaires de l'autre officine l'eurent rachetée. Malheureusement, la seule structure présente à ce jour n'est pas en capacité d'absorber l'affluence des clients, enrichie par la venue de résidents de communes périphériques. De plus, sa situation- places de parking inexistantes, accessibilité difficile -contraint les personnes à se reporter vers d'autres pharmacies, situées par exemple dans des centres commerciaux. Pour la seconde commune, le maire a dû faire preuve d'un acharnement exemplaire, en mobilisant la justice pour qu'elle donne raison à un couple proposant un projet de reprise pérenne de l'officine et non à ceux qui, disposant d'un capital certes plus élevé, souhaitaient la fermer. Face à de telles pratiques, les élus locaux, principaux acteurs de la dynamique de leur territoire, demeurent désemparés. La situation des habitants est elle aussi fragilisée. Ainsi, comment peut-on accepter l'acquisition d'une officine en vue d'une cessation définitive de son activité quand, dans le même temps, la population de la commune augmente, que la présence de professionnels médicaux est assurée- installation de plusieurs médecins généralistes, construction d'une maison médicale -et qu'un projet de reprise existe Le droit en vigueur ne permet pas, en pratique, de répondre à cette problématique. C'est pourquoi cet amendement tend à mieux encadrer juridiquement ces procédés. Quel est l'avis de la commission ? de la commission ? Cet amendement vise sans doute à répondre à des difficultés concrètes qui ont pu être constatées, mais ces dispositions ne paraissent pas devoir figurer dans la loi. Sur ce sujet, qui a fait l'objet d'une ordonnance récente, nous souhaitons avoir l'avis du Gouvernement.

L'article du code de la santé publique visé par votre amendement concerne les cessions d'officine réalisées dans le cadre d'une opération de restructuration permettant de répondre à la problématique des communes en surdensité officinale. Ainsi, les officines en difficulté du fait d'une offre surabondante en un même lieu peuvent espérer obtenir un financement de la part des pharmacies voisines en échange de leur fermeture. Il s'agit de transactions d'ordre privé, sur lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé est consulté pour avis.

à Mme Élisabeth Doineau. Les ressources hospitalières peuvent parfois constituer un point d'appui précieux pour renforcer l'accès aux soins. C'est notamment le cas dans certains territoires dénués de ressources et d'initiatives libérales. nous sommes l'assemblée des territoires, je vais citer deux exemples- mais je pourrais en citer beaucoup d'autres. En Lot-et-Garonne, le déploiement de consultations avancées entre sites hospitaliers permet de renforcer l'offre spécialisée de proximité. Également, la projection de ressources hospitalières dans des structures en ambulatoire, sur le modèle du centre médical de la Grande-Garenne, à Angoulême, permet de garantir, grâce à l'attractivité du statut salarié hospitalier, l'accès à des consultations médicales dans certains territoires dépourvus de ressources libérales. Ce type d'action permet à l'établissement de santé d'affirmer son rôle de pivot dans l'organisation des soins sur le territoire. Pourtant, elles doivent au préalable susciter l'adhésion des professionnels et peinent par ailleurs à trouver un modèle économique et organisationnel stable. Les actes tarifés suffisent rarement à couvrir l'ensemble des dépenses de fonctionnement et d'organisation. Les retours sur investissement, comme la diminution des passages aux urgences, du recours aux transports sanitaires, sont difficilement chiffrables, mais ils sont réels. Cette situation peut donc s'avérer très problématique dans un contexte budgétaire contraint pour les hôpitaux. L'amendement que je vous soumets vise à valoriser la responsabilité territoriale des établissements de santé, à l'heure où le Gouvernement entend revaloriser les soins de proximité dispensés par les établissements de santé. d'objectifs et de moyens, ou CPOM, des établissements de santé serait un levier puissant pour mieux reconnaître les démarches de ce type et, surtout, les valoriser. La création des hôpitaux de proximité est l'occasion de conduire cette réflexion. Enfin, la création d'un financement dédié à la responsabilité territoriale sur critères ou sur projet permettrait d'assurer l'équilibre financier des projets favorisant l'accès territorial aux soins dans les zones sous-denses. Quel est l'avis de la commission ?

pour développer des modes d'intervention en direction des territoires les plus isolés, comme la télémédecine ou des consultations avancées. La commission émet un avis favorable. Quel est

est déjà satisfait. Il est prévu que les contrats fixent les éléments relatifs aux missions de soins ou de santé publique spécifiques assignées à l'établissement de santé, de même que les actions de coopération engagées. Il nous semble donc que le cadre législatif actuel est suffisant pour rendre compte des actions engagées au titre de la réduction des inégalités territoriales de santé- on est bien dans le cadre de la santé publique

pour faciliter l'accompagnement et la prise en charge des patients en situation complexe. Ils aident les professionnels à trouver des solutions concrètes afin d'éviter les ruptures de parcours et de prévenir les hospitalisations inutiles ou évitables. Pour autant, les territoires d'intervention de ces dispositifs ne sont pas toujours harmonisés au niveau local. Cet amendement vise donc à mieux structurer l'offre de santé de proximité et d'appui à la coordination. Il tend à mettre en place un cadre simplifié pour que les acteurs puissent déterminer eux-mêmes les modalités d'organisation de ce dispositif d'appui à la coordination des parcours complexes, en tenant compte des réalités locales, des besoins de la population et de leurs propres besoins. L'amendement prévoit donc de maintenir les dispositifs et les missions d'expertise à vocation régionale, par exemple les réseaux régionaux en cancérologie ou en périnatalité. De plus, il a pour objet de permettre aux conseils départementaux qui le souhaitent d'inclure les centres locaux d'information et de coordination dans le périmètre des dispositifs d'appui à la coordination afin de réunir l'ensemble des services aux usagers et aidants, avec l'appui des professionnels, chaque fois que cela est possible et pertinent. Je ne doute pas que cet amendement de simplification retiendra l'attention et séduira mon collègue René-Paul ! Quel est l'avis de la commission ?

d'une dispersion des outils d'appui à la coordination des parcours complexes. Une logique de guichet unique paraît souhaitable, de même qu'une meilleure articulation avec les CPTS, qui jouent également un rôle de coordination de parcours du patient. C'est la raison pour laquelle la commission émet un

Aussi, la prévention, notamment celle des pathologies, constitue un enjeu considérable. Dans cette perspective, la mise à disposition d'informations ne saurait constituer l'unique moyen pour répondre à cet objectif. La prévention menée au niveau local, par exemple, doit s'appuyer sur des équipes pluridisciplinaires. Les acteurs de l'éducation thérapeutique et les professionnels de la relation d'aide sont appelés à trouver leur place. Inciter les personnes à optimiser leurs propres ressources doit être pris en compte dans la transformation du système de santé.

lesquelles cet amendement vise à mieux encadrer la présence, au sein des centres et maisons de santé, d'autres professionnels, tels que les hypnothérapeutes et les psychologues. Quel

Pour les autres personnels, il faut être vigilant dès lors que les contours de la profession ne sont toujours pas bien définis. S'agissant des hypnothérapeutes visés dans l'objet de l'amendement, l'évolution proposée ne paraît pas, en l'occurrence, la mieux adaptée en vue d'amorcer une reconnaissance de cette profession.

est réservée aux professionnels médicaux. La profession d'hypnothérapeute n'existe donc pas en tant que telle et les personnes qui revendiquent ce titre n'ont ni la formation ni le niveau des professionnels de santé. Votre amendement expose ainsi au risque d'introduire systématiquement dans les centres et maisons de santé des pratiques non conventionnelles et non éprouvées scientifiquement. La protection de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients étant un enjeu majeur, je ne peux être que défavorable à cet amendement.

Le morcellement du système de santé actuel rend difficiles la définition et la mise en cohérence d'une véritable politique de santé. Les multiples strates de la gouvernance rendent le système opaque pour les organisations, les élus, les professionnels et les usagers. Lors des auditions menées en amont de ce projet de loi, notamment sur l'organisation du système de soins, dans le cadre de la mission dont ma collègue Véronique Guillotin était corapporteur, nous avons pu mesurer les difficultés rencontrées par tous les acteurs de la santé en raison de cette opacité, dont beaucoup se sont plaints.

je vais peut-être réussir ! C'est le dernier ! À ce jour, les infirmiers peuvent effectuer certaines vaccinations sans prescription médicale. Ils peuvent aussi renouveler, sous certaines conditions, les prescriptions datant de moins d'un an de médicaments contraceptifs oraux. Le présent amendement a pour objet d'élargir ce droit. Ainsi, il vise à permettre à ces professionnels, dans un cadre sécurisé, de renouveler certaines prescriptions de médicaments, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Enfin, une telle mesure permettrait de réduire l'impact de la désertification médicale sur les territoires ruraux, les coûts de transports pour les citoyens- carburant, tickets de transport ... -, et représenterait une source d'économies pour l'assurance maladie en évitant une consultation du médecin. Quel

l'avis du Gouvernement ? De manière générale, vous le savez, les infirmiers ne sont pas autorisés à prescrire des médicaments compte tenu des responsabilités et des incidences importantes que cela implique et au regard des compétences acquises au cours de leur formation.

d'adapter certains traitements, à condition qu'il intervienne dans le cadre d'un exercice coordonné et sur une liste de traitements fixée après avis de la HAS. Par ailleurs, le droit de prescription a été reconnu pour les infirmiers de pratique avancée qui devraient sortir des écoles et des masters l'année prochaine. Ces infirmiers de pratique avancée se voient déléguer, sous certaines conditions, des compétences relevant du champ médical. Dans ce cadre,

Cet amendement vise à étendre les compétences des infirmiers afin de répondre aux besoins des patients et aux nouveaux enjeux de santé publique, en leur permettant de prescrire certains médicaments. Alors que le projet de loi vise à « transformer le système de santé », il paraît logique d'apporter des modifications de fond attendues par les professionnels de santé et les patients en assouplissant le cadre légal existant de la prescription. Cette mesure de bon sens, qui s'adresse essentiellement aux infirmiers libéraux, permettra un meilleur suivi des pathologies diagnostiquées par les médecins et une meilleure prise en charge de la douleur. L'arrêté ministériel prévu par l'amendement devra, en amont de sa publication, permettre de consulter l'ensemble des sociétés savantes concernées afin de déterminer une liste acceptée par les professionnels de santé qui sera, bien entendu, limitée aux besoins exprimés dans les territoires et transmis par les ordres. La Cour des comptes formule la même recommandation pour le cadre hospitalier : déléguer plus d'actes afin de répondre aux problématiques de démographie médicale.

les éléments qui viennent d'être présentés par ma collègue Dominique Estrosi Sassone, me contenant de souligner deux points. Dans cette réorganisation que nous envisageons de la médecine de ville et de la médecine ambulatoire, deux catégories d'acteurs sont particulièrement intéressantes : les pharmaciens et les infirmiers Les pharmacies constituent aujourd'hui un réseau qui continue de mailler les territoires, en particulier les zones rurales. zones rurales. Les infirmiers sont des acteurs de santé qui se rendent au domicile des patients et sont donc au contact de leur vie quotidienne.

vise à assouplir le cadre légal d'exercice des infirmiers. Ainsi, l'infirmier pourra, par exemple, prescrire les examens de contrôle du patient diabétique dont il assure le suivi. La dépose des dispositifs médicaux que les infirmiers prescrivent déjà serait également facilitée. Cette mesure sera source de simplification pour les professionnels autant que pour les patients

de la commission ? Ces amendements étendent de manière un peu large- trop large ! -le pouvoir de prescription de l'infirmier, y compris en dehors d'un exercice dans le cadre d'une prescription médicale.

tel que le paracétamol, par exemple. En effet, l'article 7 tend à autoriser les infirmiers et infirmières à prescrire des dispositifs médicaux qui existent en vente libre. Les antalgiques de palier I sont également déjà disponibles en vente libre et pourraient donc être prescrits prescrits par les infirmiers et infirmières, ce que demande la FNESI, la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers. Il serait d'ailleurs relativement ironique, pour ne pas dire ubuesque, que des patients puissent s'en procurer dans des supermarchés, alors que des professionnels de santé qui ont suivi un enseignement de la pharmacologie pendant trois ans ne pourraient pas les prescrire ! Rappelons que l'acte de prescription permet également de sensibiliser le patient sur son usage, sur les dosages et les dangers éventuels ou les effets indésirables. Trop souvent, ces médicaments apparaissent presque anodins et les patients ignorent leur toxicité. Ouvrir aujourd'hui ce médicament à la prescription des infirmiers et infirmières permettrait permettrait donc de sécuriser son utilisation et, surtout, de faire un relais d'orientation du patient vers le médecin pour éviter des retards de diagnostic de certaines pathologies, parfois camouflées par une prise d'antalgiques non encadrée.

Enfin, cet élargissement des compétences de ces professionnels de santé correspond, me semble-t-il, à la philosophie de ce que vous souhaitez mettre en oeuvre, madame la ministre, notamment par cette loi ou, plus largement, avec votre plan Ma santé 2022. Notre amendement va tout à fait dans

libre ! Sans ordonnance, soit ! Vous avez raison, il faut employer les bons termes et je remercie mes collègues pharmaciennes et pharmaciens

La Haute Autorité de santé a affirmé, dans son avis du 15 janvier dernier, « qu'une extension de la prescription [des tire-laits] aux infirmières puéricultrices pourrait être envisagée dans la mesure où elles participent déjà à l'accompagnement à l'allaitement ». l'allaitement ». Elles n'ont pas ce droit de prescription ouvrant au remboursement. En effet, l'article R. 4311-13 du code de la santé publique précise que l'infirmière titulaire du diplôme d'État de puéricultrice dispense en priorité les actes de surveillance du régime alimentaire du nourrisson. Le diplôme d'État de puéricultrice est délivré aux titulaires d'un diplôme d'infirmier ou de sage-femme qui ont validé une formation spécifique. Aujourd'hui, parmi eux, seules les sages-femmes ont l'autorisation de prescrire des tire-laits. Il apparaît donc justifié de faire évoluer par la loi la possibilité de prescription de dispositifs de soutien à l'allaitement tels que les tire-laits par les puéricultrices, puis de définir précisément les dispositifs concernés dans le cadre ministériel. Les deux

Les centres de protection maternelle et infantile, ou PMI, les parents, les puéricultrices prodiguent beaucoup de conseils, notamment au sujet de l'alimentation du bébé. Il semble donc logique de leur permettre de prescrire les dispositifs de soutien à l'allaitement. les actes dispensés en priorité par une infirmière titulaire du diplôme d'État de puéricultrice figure « la surveillance du régime alimentaire du nourrisson Madame la ministre, vous avez répondu à nos collègues députés qu'il existe moins d'une centaine de puéricultrices libérales en France et que cette disposition ne facilite que faiblement l'accès aux soins.

de prescrire des dispositifs médicaux lorsqu'ils agissent sur prescription médicale. La modification souhaitée pourrait être résolue par une adaptation de l'arrêté ministériel fixant la liste des dispositifs médicaux concernés.

n'est absolument pas l'unique vecteur de cette amélioration de l'accompagnement des femmes et de leurs enfants. Deux rapports parlementaires relatifs aux missions des centres de PMI et au parcours de santé des enfants jusqu'à 6 ans sont à l'origine d'une feuille de route sur les mille premiers jours des enfants

qu'il faut étudier les possibilités de faire évoluer plus largement le champ des compétences des infirmières puéricultrices dans la prise en charge de l'enfant dès les premières années de la vie. Pour ces raisons et dans l'attente de la réalisation de tous ces travaux qui devront impliquer l'ensemble des professionnels

en affrontement entre ces différentes professions, qui viendraient se disputer les actes à réaliser. Dès lors, il faut que ces professions participent aux discussions sur la délimitation de leurs compétences et de leurs responsabilités.

d'intérêt ou de respect pour la profession d'infirmière puéricultrice, mais pour que le nouveau système de soins se construise de façon participative et régulée, et non dans la confusion et la concurrence.

Monsieur Vaspart,

pourra, à la suite de cette première consultation, soit prendre en charge le patient, soit le réorienter vers son médecin traitant. Cela permettra de mieux traiter la petite traumatologie telle qu'entorses ou lumbagos et d'être plus efficace dans la prise en charge.

du droit de prescription. Dans un objectif de pertinence des soins, il a paru utile à la commission de maintenir le médecin traitant comme un pivot de la prise en charge des patients et de la régulation de l'accès à ces soins, dont la croissance est particulièrement dynamique.

En abordant la pratique de l'ostéopathie dans les zones sous-denses, nous entendons démontrer que de telles initiatives devraient être envisagées, en liaison avec une structure ayant autorité. Cela impliquerait de saisir le conseil départemental de l'ordre des médecins, faute de conseil de l'ordre des ostéopathes. La solution proposée n'est pas des plus orthodoxes, puisqu'elle revient à demander au Conseil de l'ordre des médecins de se prononcer sur la demande d'un non-médecin. En l'état actuel du droit, aucune solution orthodoxe ne permet de sécuriser les initiatives des ostéopathes. Seule la création d'un conseil de l'ordre des ostéopathes permettrait de remédier à cet angle mort de notre législation.

Je me réjouis que la commission des affaires sociales ait adopté cette disposition, qui conforte et renforce la dimension profondément humaine de l'engagement des infirmiers. des infirmiers. Nous venons de passer deux jours à déplorer les méfaits de la désertification médicale qui gangrène nos territoires. Aujourd'hui, la notion de « médecin de famille », ce médecin qui guérissait nos plaies et qui pansait nos âmes, est derrière nous. Les paradigmes ont totalement changé. Alors, qui reste-t-il sur le terrain ? Aujourd'hui, 116 000 infirmiers exercent, pour 90 % de leur temps, à domicile. Chaque jour, 700 000 patients en situation de dépendance

lien indispensable et bienveillant qui rend cette profession si humaine. Par conséquent, il me semble que ce rôle de coordination est fondamental.

d'infirmier est amenée à jouer un rôle central dans la transformation de l'organisation de notre système de soins, au regard de l'enjeu de santé publique considérable que représente la transition démographique en cours. Dans le cadre du premier recours, de la collaboration avec le médecin traitant dans la prise en charge des patients âgés et chroniques, et de leur rôle en santé publique, les infirmiers doivent voir leurs missions évoluer. À cet égard, nous accueillons comme un signal positif le travail que vous engagez, madame la ministre, sur le développement des pratiques avancées. Alors que le programme Santé 21 de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Europe consacre le concept d'infirmière « de famille » ou d'« infirmier référent » et que beaucoup de nos voisins européens l'ont déployé,

Je ne vois pas en quoi la désignation d'un infirmier référent remettrait en cause la coordination déjà assurée par les CPTS et détournerait les patients de l'équipe de soins. En outre, la dénomination de « référent

Au même titre que les mesures de redistribution de tâches dont nous discutons, on remarque que les potentiels de certaines professions paramédicales demeurent largement sous-exploités. Nous ne pouvons que le regretter. L'amendement

présent article prévoit que le médecin traitant, le pharmacien correspondant et l'infirmier référent soient signataires d'un même projet de santé d'exercice coordonné. C'est confondre,

à apporter une dérogation à l'interdiction du partage d'honoraires qui porte le nom assez peu élégant de « compérage ». En effet, aujourd'hui, l'activité des soins infirmiers à domicile relève le plus souvent d'une rémunération forfaitaire, et non d'un paiement à l'acte. Or, du fait de l'obligation déontologique de continuité des soins édictée par l'article R. 4312-12

Aussi, les infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant à ce titre une rémunération forfaitaire par patient pourraient ne pas être soumis à l'interdiction de partage d'honoraires au sens du code.

Les médecins, les pharmaciens et les autres professionnels de santé sur un même territoire doivent pouvoir coopérer facilement, sans passer par des voies dérogatoires, et ce afin de faciliter l'accès aux soins des patients. Quel est l'avis de la commission

la portée de ce dispositif dont la montée en charge sera évidemment progressive, puisqu'elle devra s'appuyer sur des protocoles, ou « arbres de décisions », entre médecins et pharmaciens. Laissons les professionnels se saisir de cette possibilité qui leur est ouverte. Je vous demande donc de bien vouloir retirer

Élisabeth Doineau. L'article 7 étend la compétence des pharmaciens en leur permettant, dans le cadre de protocoles inscrits dans un exercice coordonné, de délivrer des médicaments figurant sur une liste fixée par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de santé et sur la base de protocoles définis par elle. Le présent amendement vise à sécuriser cette disposition et à la rendre plus opérationnelle. lieu, de mentionner que la liste fixée par arrêté précise également les pathologies auxquelles sont associés les médicaments pour lesquels la délivrance par les pharmaciens est autorisée. En effet, un même médicament peut être utilisé pour plusieurs pathologies.

de loi, qui permet la rédaction de protocoles nationaux par les équipes s'inscrivant dans un exercice coordonné, puis leur autorisation par arrêté ministériel après avis de la HAS. Je précise que cet amendement correspond aux préconisations de la Haute Autorité de santé elle-même.

est ainsi libellé : La parole est à M. Max Brisson. Cet amendement vise à étendre, à titre expérimental, la vente de médicaments non soumis à prescription médicale dans les établissements où une personne est titulaire d'un diplôme français d'État de docteur en pharmacie ou de pharmacien.

la vente en ligne ne permet pas aux patients de recevoir de conseils adaptés, délivrés par des docteurs pharmacie. En outre, elle a un impact environnemental supérieur de 7 % à celui du commerce physique. la maîtrise de l'énergie, un achat en ligne équivaudrait à l'émission de 12 grammes de CO2, soit celle d'un trajet d'un kilomètre en voiture. Enfin, cette requête a été défendue par de nombreux acteurs depuis plusieurs années

depuis 2012. Pour rappel, le Sénat a déjà approuvé la mise en vente de tests de grossesse et de produits pour lentilles de contact en dehors des pharmacies, permettant un gain de pouvoir d'achat important pour les Français. Il faut continuer dans cette voie ! Quel est l'avis de la commission

Elle devrait par ailleurs se faire en concertation étroite avec les représentants de la profession, car elle remettrait en question les strictes règles démographiques qui s'appliquent pour l'installation des officines.

et des statistiques du ministère de la santé, la Drees, a pointé une surmortalité importante chez les personnes hospitalisées pour une fracture du col du fémur, principale conséquence de la fragilité osseuse des patients ostéoporotiques. Pourtant, une baisse de la prise en charge dans ce domaine a été constatée depuis 2011, ce qui se caractérise par une hausse des hospitalisations pour fracture ainsi qu'une baisse du nombre d'ostéodensitométries réalisées. Aussi proposons-nous, dans le cadre de l'amélioration des parcours de soins pour l'ostéoporose présentée au sein du plan Ma santé 2022 et des nouvelles missions du pharmacien d'officine, de permettre à ce dernier de proposer un questionnaire de dépistage de l'ostéoporose aux femmes de plus de 50 ans,

Cet amendement vise à développer les compétences des pharmaciens en les autorisant à contrôler la tension artérielle, ainsi qu'à délivrer des médicaments pour une cystite et à pratiquer préalablement un examen cytobactériologique des urines, Bien sûr, les pharmaciens devront, dans le cadre d'un protocole, communiquer les résultats de ces examens au médecin traitant et les inscrire dans le DMP, le dossier médical partagé du patient. Les pharmaciens

amendement a le même objet que l'article 7 , qui permet au pharmacien de délivrer sans prescription médicale préalable des produits de santé de premier recours pour des situations simples,

Si l'on peut se réjouir de cette baisse significative, il faut toutefois garder à l'esprit que le tabagisme reste, malheureusement, la première cause de décès évitable en France. Afin de renforcer la lutte contre le tabagisme, nous proposons, à travers cet amendement, de faciliter l'accès aux substituts nicotiniques, qui peuvent être actuellement prescrits par les médecins, les sages-femmes et divers autres professionnels de santé, en autorisant les pharmaciens d'officine à prescrire ces substituts, ce qui faciliterait le parcours d'aide au sevrage tabagique. Je sais toutefois, madame la ministre, que vous considérez que ce n'est pas une bonne mesure que de prévoir que le conseiller et le prescripteur soit la même personne que le vendeur. Je rappellerai simplement que les étudiants en pharmacie, à la fin de leur soutenance de thèse, prononcent le serment de Galien : ils jurent alors d'exercer leur profession dans l'intérêt de la santé publique et avec conscience, et de respecter, non seulement la législation en vigueur, mais aussi les règles de l'honneur, de la probité et du désintéressement.

Cependant, il faut parfois attendre plusieurs jours pour avoir un rendez-vous chez son médecin et obtenir une ordonnance de substituts nicotiniques. Pour rencontrer un médecin tabacologue, les délais de rendez-vous sont de trois ou quatre semaines. Cela peut freiner les patients dans leur volonté d'arrêter de fumer. Aussi, afin de répondre efficacement et rapidement à la décision du patient, le pharmacien d'officine doit pouvoir prendre l'initiative d'un traitement de substituts nicotiniques pris en charge par l'assurance maladie. Par ailleurs, la convention pharmaceutique prévoit de travailler avec les syndicats de pharmaciens d'officine pour définir un dispositif de lutte contre le tabagisme. Dans le cadre de cette stratégie conventionnelle de prévention, le pharmacien d'officine accompagnera le patient pendant toute sa période de sevrage tabagique par la mise en place d'entretiens motivationnels, un accompagnement médical n'étant pas indispensable dans ce cas. En outre, cette autorisation de prescrire des substituts nicotiniques est déjà ouverte pour les dentistes, les sages-femmes, les infirmières et les kinésithérapeutes, mais pas pour les pharmaciens, alors même qu'ils se trouvent régulièrement en lien avec ces patients dans le cadre de pathologies associées ou autres. De plus, leur consommation ne se fera, étant donné leur nature, que selon leur strict besoin. On n'imagine pas quelqu'un se mettre un patch nicotinique s'il n'en a pas besoin ! Le tabac a fait 75 000 morts en France en 2015, soit plus d'un décès sur huit. Il serait regrettable de priver le patient de la chance de se faire prescrire des substituts nicotiniques lors d'entretiens avec son pharmacien. Il paraît donc naturel de laisser aux pharmaciens d'officine la possibilité de prescrire des substituts nicotiniques, afin d'améliorer les taux

de la commission ? Les substituts nicotiniques peuvent déjà être prescrits par les sages-femmes, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes, au-delà des seuls médecins et médecins du travail. Faut-il étendre ce droit de prescription aux pharmaciens d'officine ?

À l'heure actuelle, conformément à l'article L. 6211-1 du code de la santé publique, les prélèvements d'anatomo-cytopathologie, bien que cotés à la nomenclature des actes de biologie médicale, restent de la compétence des médecins. Ainsi, si les biologistes médicaux pharmaciens sont formés et réalisent quotidiennement des prélèvements vaginaux en vue d'examens cytologiques, bactériologiques ou virologiques, ils sont contraints de renvoyer les patientes vers des médecins pour la réalisation de frottis cervico-vaginaux à des fins de dépistage du cancer du col de l'utérus, alors qu'il s'agit de la même technique de prélèvement. Permettre aux biologistes médicaux pharmaciens, qui représentent 75 % des biologistes médicaux, 75 % des biologistes médicaux, d'effectuer ce type de prélèvement faciliterait l'accès au dépistage du cancer du col de l'utérus.

surveiller beaucoup plus régulièrement.

professionnels capables d'accompagner globalement la femme dans ces pathologies cancéreuses et ces pathologies féminines.

cadre du plan Cancer, nous avons voulu organiser le dépistage du cancer du col de l'utérus au même titre que le dépistage du cancer du sein et du dépistage colorectal, ce qui permet une prise en charge à 100 % par l'assurance maladie. De nombreux scénarios de dépistage ont été évalués avec des expérimentations. Il est apparu qu'un dépistage tous les trois ans qui reposait sur une lettre d'invitation envoyée à toutes les femmes dans la tranche d'âge 25-65 ans,

par la direction générale de la santé lors des expérimentations ; il n'est pas remboursé, parce que la HAS ne l'a pas validé à ce jour comme étant utile.

Hormis l'accompagnement de la réforme des études de santé et la régulation de l'offre de soins, elle a estimé que la libération de temps médical, notamment par le développement des partages de compétences, devait constituer une priorité. Plusieurs dispositions introduites à l'Assemblée nationale vont d'ailleurs dans ce sens, certaines d'entre elles ayant été supprimées par la commission des affaires sociales du Sénat, comme le renforcement des compétences des orthoptistes. durable considère que tout n'a pas été tenté pour libérer du temps médical dans nos territoires et pour utiliser au mieux les ressources médicales dont nous disposons en partageant les compétences entre professionnels de santé. Certaines professions médicales sont pourtant mieux réparties sur le territoire et bénéficient d'une démographie dynamique. C'est notamment le cas des sages-femmes, dont les effectifs ont augmenté dans une forte proportion depuis 2000- de 50 % selon la Cour des comptes. Comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, à la suite de la mise en place de mesures de régulation, la répartition territoriale des sages-femmes s'est d'ailleurs largement améliorée, selon une récente étude du ministère. Il s'agirait donc de mieux s'appuyer sur les compétences de ces professionnels de santé pour libérer du temps médical dans nos territoires. Lors des auditions que j'ai menées, il est pourtant apparu que les restrictions de compétences des sages-femmes par des listes limitatives déterminées par voie réglementaire exposaient les femmes à une double consultation, d'abord auprès de la sage-femme, d'abord auprès de la sage-femme, puis auprès du médecin. L'élargissement du droit de prescription des sages-femmes proposé par la commission constitue ainsi une solution pragmatique et de bon sens permettant de simplifier le parcours de soins de nos concitoyens. Je signale à ce sujet que le droit à la pleine prescription existe déjà pour une autre profession médicale, celle de chirurgien-dentiste. De manière pragmatique, notre commission a d'ailleurs fait évoluer la mesure qu'elle avait proposée initialement, en précisant en précisant que ce droit de prescription ne serait limité qu'aux dispositifs médicaux strictement nécessaires à l'exercice de leur profession et en renvoyant les conditions d'application de ces dispositions à un décret en Conseil d'État. Quel est l'avis de la commission ? de la commission ? On aborde ici les conditions globales d'exercice d'une profession de santé, alors que ce n'est pas l'objet du projet de loi. L'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM, sur les médicaments prescriptibles par les sages-femmes constitue par ailleurs un moyen de sécurisation pertinent. En outre, les sages-femmes peuvent déjà pratiquer tous les actes nécessaires à l'exercice de leur profession et précisés dans la partie réglementaire du code de la santé publique. Elles peuvent en pratiquer certains d'office, sans prescription, et d'autres sur prescription du médecin en cas de grossesse pathologique- dans ce cas précis, il est nécessaire d'avoir un cadre.

au cours du parcours de soins, assurer un rôle plus important et être les professionnels de premier recours lors de la grossesse, avant le déclenchement de la consultation médicale. Les recommandations de la Cour d'un point de vue tant médical que budgétaire, visaient deux objectifs : d'une part, mieux articuler et valoriser les compétences des sages-femmes, d'autre part, réorienter leur activité vers des actes à plus forte responsabilité, notamment le suivi postnatal. Outre un ensemble de missions déterminées pour le suivi médical de la grossesse, puis du nouveau-né, il est précisé que la sage-femme ne peut pas remplacer les médecins référents, mais que sa fonction permet permet de contribuer à l'offre de soins sur le territoire et de répondre ainsi à l'angoisse de certains parents, notamment lors des premières semaines de l'enfant, évitant de déclencher peut-être une consultation pédiatrique pédiatrique ou gynécologique, qu'elle soit en ville ou en établissement hospitalier, ce qui représente aussi une économie pour la sécurité sociale.

par la même personne. Si le suivi est réalisé par un groupe de professionnels de santé, une personne " référente " dans ce groupe facilite la coordination et l'organisation des soins et leur articulation avec le secteur social et les réseaux d'aide et de soutien. » Aucune différence n'a été relevée, que le praticien soit un obstétricien, un gynécologue,

à Mme Laurence Cohen. Avant d'aborder à l'article suivant la définition des équipes de soins spécialisées, nous proposons nous aussi de reconnaître la place des sages-femmes dans les équipes de soins primaires. En effet, les actions de dépistage, de prévention et de diagnostic des pathologies effectuées par les sages-femmes font d'elles des praticiennes de premier recours en soins primaires pour la santé des femmes. Ces professionnelles sont donc au coeur du dispositif permettant à la patiente d'être au centre du parcours de santé. Cette place dans le système de santé français nécessite, selon nous, d'être clairement inscrite dans la loi. Un parcours de santé se définit comme la trajectoire globale des patients dans leur territoire, une attention particulière étant portée à la personne et à ses choix. Le parcours de santé des femmes est l'organisation d'une prise en charge globale et continue, au plus proche de leur lieu de vie ou de travail. La lisibilité, l'accessibilité et la fluidité du parcours de santé s'appuient sur la qualité de l'information, des conditions d'accueil et d'accompagnement de la femme tout au long de sa vie. Tous ces arguments plaident en faveur de la reconnaissance des sages-femmes dans les équipes de soins primaires, conformément à la philosophie du plan Ma santé 2022, et de l'élargissement des compétences de certaines professionnelles, s'agissant plus spécifiquement de la santé des femmes.

pour le suivi gynécologique, contraceptif et préventif, mais aussi pour le suivi postnatal. On peut néanmoins s'interroger sur la portée réelle de l'inscription dans la loi de la notion de sage-femme « référente En effet, la revalorisation des actes à forte responsabilité médicale pratiqués par les sages-femmes, en l'espèce les consultations, les accouchements et le suivi postnatal, suppose la révision de la nomenclature de ces actes

que tous les professionnels de santé concourent à l'offre de soins de premier recours. Les sages-femmes en font logiquement partie. Par ailleurs, la partie réglementaire du code de la santé publique- c'est l'article R. 4127-318 -détaille précisément les responsabilités des sages-femmes,

Lubin. Madame la ministre, huit maisons de naissance ont été ouvertes à la suite de la loi du 6 décembre 2013 autorisant leur expérimentation et du décret du 30 juillet 2015 précisant les conditions de cette L'arrêté du 23 novembre 2015 a marqué le début de la période d'expérimentation de cinq ans. Ces maisons offrent un accompagnement des naissances plus personnalisé et plus intime,

En cas de nécessité, les transferts de la mère ou du nouveau-né se font vers l'établissement de santé partenaire. Les rapports d'évaluation réalisés à ce stade de l'expérimentation font déjà état de la grande satisfaction des parents, des sages-femmes et des équipes hospitalières partenaires des maisons de naissance, mais également de la sécurité et des bons résultats en termes de santé de ces structures. Cet amendement vise donc à introduire, de manière pérenne, la définition des maisons de naissance dans le code de la santé publique, et ce pour plusieurs raisons. Une telle offre de suivi permet aux professionnels de disposer de plus de temps avec les futurs parents tout au long de la grossesse et au moment de l'accouchement, grâce au ratio une femme pour une sage-femme, ce qui s'inscrit tout à fait dans la stratégie Ma santé 2022 mise en oeuvre par le Gouvernement. La pratique des maisons de naissance est particulièrement économique. En outre, il a été démontré qu'une moindre médicalisation et le respect de l'intimité tendent à faciliter l'accouchement et à favoriser l'établissement du lien parent-enfant. avantages connus expliquent la prévalence de ce type de lieux de naissance dans de nombreux pays européens, notamment dans les pays scandinaves, où 40 % des accouchements ont lieu dans de telles

Enfin, l'anticipation de la suite de l'expérimentation permettrait d'éviter le risque de rupture dans la prise en charge des parents qui seront accueillis durant l'année à venir.

L'expérimentation des maisons de naissance a été lancée en 2015 pour une durée de cinq ans. Au total, neuf maisons de naissance sont en cours d'expérimentation. Il est préférable, à notre avis, d'attendre l'évaluation complète

madame la ministre,

qui sont surchargés, sachant en outre que les délais d'attente pour obtenir un rendez-vous sont longs, notamment dans les territoires ruraux, mais aussi dans les quartiers défavorisés ou sous-dotés.

aux infirmiers de pratiquer l'ensemble des vaccinations de l'adulte sans prescription médicale, à l'exception de la première injection, alors que leurs compétences vaccinales sont aujourd'hui encadrées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Haute Autorité de santé. simplement, la vaccination antigrippale. Pour rappel, depuis un décret du 25 septembre 2018, les infirmiers sont autorisés à pratiquer les primo-injections de la vaccination antigrippale, ce qui représente un progrès.

Par ailleurs, le Gouvernement a saisi la Haute Autorité de santé de l'extension des compétences vaccinales des infirmiers, des pharmaciens et des sages-femmes. Il est préférable d'attendre cet avis pour envisager un dispositif plus global de renforcement des opportunités vaccinales. En attendant, la commission demande le retrait de ces amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

n° 74 rectifié. Le présent amendement vise à étendre aux 4 000 biologistes médicaux la possibilité d'administrer, sans prescription médicale, le vaccin contre la grippe saisonnière. Cela permettrait d'atteindre rapidement le taux de 75 % de couverture vaccinale fixé par la Haute Autorité de santé. Contrairement aux pharmaciens d'officine, les biologistes, qui disposent de personnels qualifiés et habilités, ayant l'expérience du prélèvement, n'auront besoin d'aucune formation préalable. Ils bénéficient d'infrastructures sanitaires, dotées de moyens informatiques et technologiques modernes. L'ensemble est régi par un système d'assurance qualité couvrant l'ensemble des processus au sein du laboratoire. Les horaires d'ouverture sont ceux des commerces. Aucune autre structure médicale non hospitalière n'offre autant de garanties pour la prise en charge médicalisée des vaccinations, mais aussi des dépistages, de la prévention et du suivi des patients chroniques.

les biologistes peuvent contribuer à l'amélioration du dispositif de prévention des épidémies grippales hivernales. Il serait dommage de se priver de leurs compétences, de leurs moyens humains et logistiques.

santé a été sollicitée en début d'année par le Gouvernement sur la question de l'extension des compétences vaccinales à d'autres vaccins et à d'autres professions de santé. Il a semblé à la commission qu'il était préférable de ne pas devancer cet avis et d'en attendre les conclusions. La commission demande donc le retrait

La commission des affaires sociales considère que l'organisation de la filière visuelle, caractérisée par des difficultés croissantes d'accès aux soins d'ophtalmologie dans plusieurs régions, doit impérativement être clarifiée. Il convient en particulier de mieux préciser les compétences respectives des différents métiers- ophtalmologiste, orthoptiste, opticien-lunettier, optométriste -et d'adapter le cas échéant leur formation. Il ne lui a donc pas semblé opportun d'adopter une nouvelle mesure ponctuelle, dont l'efficacité et la cohérence avec la réorganisation d'ensemble de la filière ne sont pas démontrées. Pour ces raisons, elle a supprimé l'article 7 C. Logiquement, elle émet un

: La parole est à Mme Chantal Deseyne. Cet amendement vise à permettre aux opticiens d'effectuer les actes préalables au bilan visuel tels que la mesure de la pression intra-oculaire ou la rétinographie. Actuellement, ils ne peuvent le faire faute d'une autorisation pour utiliser les appareils nécessaires à ces mesures, l'interprétation, le diagnostic et la prescription restant de la seule compétence de l'ophtalmologiste. Cet amendement permettrait de dégager du temps médical, particulièrement dans les zones sous-dotées, où il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous. Plusieurs projets d'expérimentation sont actuellement bloqués faute, pour l'opticien, de pouvoir utiliser ces appareils.

30 % des parents sont aujourd'hui confrontés à des problèmes de vue pour leurs enfants, 10 % des enfants de moins de 5 ans souffrent de problèmes de vue, 13 % des enfants de 4 ans à 10 ans sont atteints de myopie, contre 10 %, semble-t-il, en 2016. Enfin, 38 % des salariés de plus de 50 ans déclarent avoir des difficultés

Le rôle de ces professionnels au sein de la filière visuelle doit impérativement être clarifié. Toutefois, les extensions de compétences en faveur des opticiens autorisées depuis 2007 ont eu jusqu'à présent des effets marginaux. Ainsi, la délivrance d'équipements d'optique médicale continue à reposer pour l'essentiel sur les ophtalmologistes. En outre, une telle clarification ne peut s'opérer qu'en travaillant sur la complémentarité entre les différents acteurs de la filière, y compris les orthoptistes. La commission des affaires sociales, en cohérence avec sa position sur l'article 7 C concernant les orthoptistes, qu'elle a supprimé, attend donc une clarification d'ensemble de la filière visuelle, et non de nouvelles mesures ponctuelles. L'amendement n° 115 rectifié prévoit plus particulièrement de mettre à jour les actes pouvant être réalisés par les opticiens-lunetiers et les équipements pouvant être utilisés par cette profession. Les dispositions proposées ne relèvent pas toutes du domaine de la loi. l'article L. 4362-11 du code de la santé publique dispose notamment que « les règles d'exercice et, en tant que de besoin, d'équipement » de la profession sont déterminées par décret.

Madame la ministre, l'article 7 ouvre un droit important pour les pharmaciens, celui de se substituer aux médecins dans la prescription d'un médicament en cas de rupture de stock. Cet article, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, va dans le bon sens, celui d'une meilleure répartition des tâches entre professionnels de santé, celui aussi d'une simplification de la vie de l'usager, en l'occurrence le malade.

à l'Assemblée nationale un plan d'action sur le sujet d'ici l'été, pour tenter de réduire le nombre et la durée de ces ruptures de stock et d'approvisionnement, mais aussi pour mieux nous organiser lorsqu'elles se produisent. Je souhaitais profiter de la séance publique pour le rappeler et vous dire, madame la ministre, que nous sommes disponibles pour décliner le rapport sénatorial et mettre en oeuvre ses recommandations dans le plan d'action que vous avez évoqué. L'amendement

L'information du pharmacien au prescripteur se ferait ainsi en amont de la prescription, et non en aval. Cela ne coûterait pas plus cher en termes de coordination et n'exigerait pas plus de travail, mais sécuriserait davantage une pratique complexe. Le prescripteur est en effet le professionnel

7 consiste précisément à permettre au pharmacien de ne pas avoir à obtenir préalablement l'accord du médecin prescripteur pour procéder à la substitution d'une spécialité en rupture, à condition qu'il procède à cette substitution dans le respect d'un protocole défini par l'Agence nationale de sécurité du médicament

avec les sociétés savantes représentant les prescripteurs. Dès qu'il y a une rupture de stock, l'ANSM travaille donc sur les médicaments de remplacement

le produit de substitution dans la liste des intervenants consultés préalablement à l'établissement de la recommandation établie par l'ANSM. Ils sont en effet les meilleurs connaisseurs de leurs produits et les mieux à même de contribuer à la discussion nécessaire autour des possibilités de substitution. Les laboratoires pourraient aussi avoir à procéder à des ajustements, tant sur la production que sur la logistique, qu'il est important de pouvoir anticiper. anticiper. Quel est l'avis de la commission ? La consultation des laboratoires exploitant les spécialités de substitution, voire des laboratoires dont la spécialité est en rupture d'approvisionnement, permettra d'éclairer sur les stocks disponibles de médicaments de substitution,

l'avis du Gouvernement ? La capacité d'approvisionnement d'une molécule de remplacement par les laboratoires suppléants est un préalable, dont l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé s'assure dans toutes les situations de rupture d'approvisionnement. Les laboratoires sont donc toujours associés pour trouver des solutions de remplacement, mais je considère que l'élaboration de la recommandation de l'ANSM quant aux produits de substitution et au protocole proposé ne relève pas de la mission des laboratoires suppléants. Cette recommandation organise organise une stratégie temporaire de prescription et de dispensation de manière indépendante et en concertation avec les associations de patients et les sociétés savantes. J'émets donc un avis défavorable. La parole est

est à Mme la ministre. Il s'agit de supprimer la possibilité donnée aux partenaires conventionnels de négocier une aide complémentaire en cas de congé maternité ou paternité pour les chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux, infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité.

Tout d'abord, l'ensemble des professionnels de santé libéraux bénéficient déjà d'une protection maternité qui représente un taux moyen de remplacement de près de 90 % du revenu des infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes. Pour les professions dont les revenus moyens sont plus bas, le taux de couverture peut atteindre 100 %. Ce régime permet ainsi aux professionnels concernés de percevoir un montant pouvant aller jusqu'à 9 600 euros durant leur congé. À titre de comparaison, le taux de remplacement moyen des revenus d'un médecin était inférieur à 60 %. C'est pourquoi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a prévu une aide financière conventionnelle complémentaire à l'indemnisation par l'assurance maladie obligatoire pour l'ensemble des médecins libéraux interrompant leur activité en cas de maternité, paternité ou adoption. Cette aide a pour objectif de favoriser l'installation des jeunes médecins, notamment dans les zones sous-denses et de renforcer l'attractivité de l'exercice libéral pour les jeunes médecins, qui s'installent plus tard et moins souvent qu'avant. L'objectif de cette aide est donc spécifique à la démographie des médecins libéraux et aux difficultés d'accès aux soins qui caractérisent cette profession. Pour toutes ces raisons, je propose un amendement de suppression de l'article

Jean-Marc Gabouty. Consulter un médecin traitant présente le double avantage d'être mieux soigné, grâce au suivi par un médecin qui connaît bien ses patients, et d'être mieux remboursé. Mais encore faut-il en avoir un ! aujourd'hui, 8,7 % des assurés de plus de 16 ans ne disposent pas d'un médecin traitant, souvent parce qu'ils n'en trouvent pas. Dans un rapport qui vous a été remis en octobre dernier, notamment par notre collègue Élisabeth Doineau, 75 caisses primaires d'assurance maladie signalent les difficultés croissantes à trouver un médecin traitant sur leur territoire. Et les personnes concernées n'ont parfois pas d'autre choix que de renoncer aux soins, parce qu'elles ne peuvent pas bénéficier d'un remboursement intégral. Aujourd'hui, il est déjà possible de se tourner vers le conciliateur de sa caisse pour tenter de débloquer la situation, mais celui-ci ne peut imposer à un médecin d'être votre médecin traitant. Aussi, nous proposons de rétablir en partie l'article 7 tel tel qu'il avait été adopté en commission à l'Assemblée nationale. Il s'agit de rendre opposable l'accès au médecin traitant pour tout assuré qui en fait la demande et effectue les démarches auprès du directeur de l'organisme gestionnaire.

La saisine du conciliateur de l'assurance maladie est déjà possible et celle du directeur de la CPAM, proposée dans ces amendements, ne changera rien à la situation.

Lors des débats parlementaires conduisant à son introduction en 2016, cet article a été complété par une notion de « coordination des soins par un médecin » dans la définition du cadre d'exercice des professionnels en pratique avancée. En réalité, le professionnel de santé en pratique avancée n'intervient pas sous la coordination d'un médecin. Il peut d'ailleurs être lui-même chargé de cette coordination. La publication des textes réglementaires relatifs à la pratique avancée étant désormais intervenue,

L'article L. 4301-1 du code de la santé publique définit l'exercice en pratique avancée des auxiliaires médicaux. Lors des débats parlementaires conduisant à son introduction en 2016, cet article a été complété par une notion de « coordination des soins par un médecin dans la définition du cadre d'exercice des professionnels en pratique avancée. En réalité, le professionnel de santé en pratique avancée n'intervient pas sous la coordination d'un médecin. Il peut d'ailleurs être lui-même chargé de cette coordination.

à délivrer des dispositifs médicaux de diagnostic destinés à réaliser des autotests de détection du VIH. En France, plus de 170 000 personnes vivent avec le VIH, près de 6 500 découvrent leur séropositivité chaque année et on estime à 30 000 le nombre de personnes porteuses du virus sans le savoir. Malgré les progrès réalisés en matière de dépistage, encore près d'un tiers des découvertes de séropositivités sont bien trop tardives. Dans une perspective de développement de l'offre de dépistage, la France a autorisé la vente en pharmacie d'autotests VIH, et c'est une bonne mesure. Ils offrent de nouvelles opportunités d'autonomie pour des personnes qui veulent faire un test en toute discrétion ou qui ont un accès plus difficile aux services de dépistage et viennent compléter l'offre En 2017, plus de 90 000 autotests ont été vendus en France, un chiffre qui ne permet malheureusement pas d'augmenter significativement le nombre de dépistages. C'est pourquoi il apparaît nécessaire de multiplier les endroits où il est possible de se procurer un autotest, notamment dans les zones à forte prévalence.

La délivrance par des infirmiers et médecins pourrait encore faciliter l'accès à ces dispositifs médicaux, mais serait une nouvelle dérogation au monopole pharmaceutique. Dans ce contexte, la commission a souhaité connaître l'avis du Gouvernement sur ce sujet.

des services spécialisés dans les grandes métropoles. La gradation des soins en trois niveaux inquiète et le recours aux ordonnances pour déterminer la liste des hôpitaux

Enfin, s'il est considéré comme un « hôpital de pointe », les services de chirurgie infantile et de gynécologie seront conservés, mais les services de premier recours seront supprimés- dans ce cas, où vont aller les patients ? Par conséquent, avec votre projet d'organisation en trois niveaux, les hôpitaux vont forcément fermer des services et l'accès aux soins se dégradera. Très bien ! La parole est à M. Bernard Jomier,

Ainsi, à rebours de la logique de surconcentration des moyens spécialisés dans les gros établissements, logique qui s'impose depuis la loi HPST comme l'évolution « naturelle » du système de santé, vous faites le choix d'amorcer un rééquilibrage en faveur de l'offre de proximité proximité qu'appelaient de leurs voeux collectivités locales, élus et citoyens. Ce rééquilibrage est conforme aux objectifs de santé publique que nous promouvons et nous ne pouvons que nous en réjouir.

Renvoyer l'intégralité de la définition de ces hôpitaux à la voie réglementaire, comme vous entendiez le faire dans le projet de loi initial, n'était pas acceptable. Vous avez bien voulu préciser votre projet, nous proposerons d'y ajouter un certain nombre d'éléments. Parmi nos propositions figure celle

me permets d'anticiper un peu le débat, mais l'article 8 ne peut pas être considéré séparément de l'article 9, par lequel vous nous demandez de vous confier un blanc-seing concernant les régimes d'autorisation des activités de soins.

l'offre de soins hospitaliers dans une logique de gradation des soins. Tout d'abord, le recours à des ordonnances témoigne de la volonté du Gouvernement d'écarter le législateur d'une question d'intérêt général, celle du maillage territorial du service public hospitalier. Il est très curieux de vouloir s'exonérer d'une discussion avec les parlementaires et les professionnels de santé sur un tel sujet. La révision de la carte hospitalière en trois niveaux laisse présager une restructuration des hôpitaux par la fermeture, au sein des petites structures hospitalières, de différents services de soins spécialisés.

Vous allez me dire que nombre de nos voisins européens fonctionnent ainsi, que c'est une vision moderne de la santé et que cette gradation des centres de soins est un gage de qualité. En réalité, votre vision est purement comptable. Cette réorganisation n'a qu'un seul but : réduire les coûts

Le 25 avril, Emmanuel Macron s'est engagé à ce qu'il n'y ait plus, d'ici à la fin du quinquennat, de nouvelles fermetures d'hôpitaux ni de maternités. Certes, vous ne fermerez pas d'établissement- le mal a déjà été fait ... -, mais vous ferez de nombre d'entre eux des coquilles vides et vous institutionnalisez une santé à deux vitesses. Très

et la biologie, mais également des missions spécialisées jusqu'à la petite chirurgie, ce qui peut rendre ces établissements attrayants aux yeux des médecins spécialistes. Il leur ouvre également la possibilité de se voir autoriser d'autres activités optionnelles, comme les soins de suite

Les conditions imposées par l'article 8 font de la médecine l'activité socle obligatoire, sans laquelle plus d'un tiers des ex-hôpitaux locaux, ceux qui ne remplissent pas cette condition, puisque cette activité leur a été enlevée, se trouveront exclus de la réforme. Dans ce cas, madame la ministre, serait-il possible d'imaginer que des établissements dépourvus d'activité de médecine pour les raisons évoquées précédemment, mais ayant une activité de soins de suite principale, ce qui ne les place pas au premier niveau de gradation, puissent postuler postuler à cette labellisation et participer de la sorte aux missions d'un hôpital de proximité, quand ils y sont prêts ? Ils sont nombreux dans cette situation, la presse s'en fait l'écho. C'est le cas en Guadeloupe du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau, dont les activités de médecine- médecine générale et hospitalisation à domicile -ont été supprimées pour les raisons que j'ai évoquées. Cet établissement public de santé vient d'être reconstruit pour plus pour plus de 85 millions d'euros d'investissement, il est situé dans un bassin de vie regroupant trois communes et comptabilisant environ 60 000 habitants et il présente toutes les garanties d'accueil, mais il souffre visiblement d'un déficit d'autorisations d'activité pour remplir l'ensemble de ses lits et rendre un service efficace à la population.

ouverte sur la ville et le secteur médico-social, et renforcer la gradation des soins ». Je souhaiterais apporter les éléments de réflexion suivants. La notion d'établissement public de santé a été introduite par la loi de réforme hospitalière du 31 juillet 1991 pour remplacer l'expression d'« hôpitaux et hospices publics

en continuité de la prise en charge des médecins de ville lors de situations de rupture nécessitant un plateau technique léger- radiologie, biologie -et/ou un hébergement sont spécifiques. Elles seront animées et gérées par des médecins généralistes en lien direct avec le secteur ambulatoire, notamment les CPTS. L'admission des patients serait facilitée par un lien direct entre leur médecin traitant et le médecin généraliste de l'établissement afin de fluidifier les parcours des patients, notamment les personnes âgées. des hôpitaux gère des situations graves ou compliquées, ils privilégient les explorations complémentaires et le recours aux plateaux techniques lourds afin d'aboutir à un diagnostic étiologique. Identifier un niveau intermédiaire spécifique, du type établissement de santé de proximité, en lieu et place de la dénomination « hôpital de proximité », permet de clarifier les niveaux de recours au sein de l'organisation du système de santé et donne de la visibilité dans le parcours de soins, en cohérence avec la gradation des niveaux de recours ambulatoires- équipe de soins et vous remercie

l'amendement n° 309. La nouvelle définition retenue par le Gouvernement va transformer les hôpitaux de proximité en véritables coquilles vides. Ils exerceront exclusivement une activité de médecine ou de soins de suite et de réadaptation.

Nous aurons ainsi des hôpitaux de seconde zone dans les territoires ruraux et périurbains et des services spécialisés et de pointe dans les métropoles et les grands pôles urbains.

ont affaibli ce qui constitue la colonne vertébrale de notre système public de santé : l'hôpital public. Nous avons vécu une succession de fermetures d'établissements, parmi lesquels de nombreuses maternités, souvent sous le prétexte de l'impossibilité d'assurer la sécurité des patientes. Aujourd'hui, c'est au nom de la pénurie médicale, qui est notamment le résultat de la mise en place d'un mortifère, que vous créez ces hôpitaux de proximité. Le maillage d'hôpitaux de proximité doit être totalement différent : il doit évidemment être maintenu, mais il doit même être développé, en s'inscrivant dans une politique d'aménagement du territoire. Nous portons avec force une autre conception de l'hôpital de proximité, qui doit être un établissement doté d'un service d'urgences, d'une maternité de niveau 1 et de services de médecine et de

en lien avec un réseau de centres de santé et la psychiatrie de secteur. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

permis de lever un certain nombre d'interrogations quant à l'impact du développement annoncé de ce modèle. Toutefois, je ne pense pas que la suppression pure et simple de cet article soit une solution raisonnable. Cela ne ferait que reporter la mise en place de la réforme, alors que la rénovation de ce statut peut aussi présenter une opportunité pour repenser la structuration des soins hospitaliers et renforcer la liaison

sincèrement qu'elles correspondent à des besoins bien identifiés, notamment par le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Nous avons été sensibles aux remarques qui ont été faites par un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale sur la nécessaire différenciation territoriale et

devons évidemment prendre le temps nécessaire pour en débattre, mais je vous demande de ne pas supprimer cet article. Je suis donc défavorable à ces amendements.

venant d'hôpitaux plus importants ou de CHU, pour leur permettre de faire des consultations avancées. Bien sûr se poseront des questions auxquelles nous n'avons pas encore eu la réponse. Je pense au financement, qui, tout naturellement, est repoussé au PLFSS,

Le travail parlementaire est donc extrêmement difficile. Pour notre part, nous allons tenter de vous accompagner en nous abstenant de voter les amendements de suppression. Nous avons présenté une dizaine d'amendements sur cet article 8. Je ne cache pas que nous sommes très dubitatifs sur la possibilité d'arriver à un accord qui soit satisfaisant sur le contenu. Je regrette encore une fois que cette procédure accélérée et la façon dont le texte a été présenté

Depuis lundi, on planche sur un texte et, quand on a une voix divergente de sa philosophie globale, rien ne passe.

qui va entraîner un éloignement des professionnels de santé. En effet, on le sait grâce aux statistiques, les professionnels de santé en libéral s'installent là où il y a une sécurité, c'est-à-dire un hôpital.

ce rapport intime avec les élus et l'ensemble des professionnels de ces territoires, pour les amener justement à comprendre comment la classification ou la labellisation pourra se faire.

Mes chers collègues, je vais lever la séance. Nous avons examiné 192 amendements au cours de la journée ; il en reste 272. La suite de